L'ordre du jour appelle l'examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. forces armées, l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux échanges de jeunes actifs

après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, sénateurs, vous le savez, les syndicats d'agglomération nouvelle, les SAN, ont été créés au début des années 80, pour organiser, structurer et financer le développement des villes nouvelles, lesquelles, dès les années 60, ont connu une expansion démographique exceptionnelle, qu'il a fallu accompagner par la production d'un nombre important de logements et la création d'équipements publics rendus nécessaires par l'accueil de nouveaux habitants, en particulier en Île-de-France, qui concentre cinq des neuf sites. Les SAN ont bénéficié d'un soutien financier de l'État multiforme, par le biais d'une facilitation de l'accès à l'emprunt, d'aide au financement des investissements ou de dotations. Rappelons que ces syndicats avaient vocation à disparaître à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement des villes nouvelles. Consécutivement à l'adoption de la loi Chevènement de 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, un statut particulier a été réservé aux SAN s'agissant du calcul de leur dotation d'intercommunalité, que cette loi a généralisé en accompagnement de l'intégration plus forte des communautés. Leur potentiel fiscal a ainsi été pondéré afin de tenir compte de leurs charges particulières, liées à un endettement important, très supérieur à la moyenne nationale, engendré par des constructions massives de logements et d'équipements conjuguées à un développement économique et une évolution des recettes fiscales progressifs, mais trop faibles pour y subvenir. Ces réalités ont donc été prises en compte dans le calcul des dotations. La modalité de calcul dérogatoire du potentiel fiscal a été maintenue dans le temps, pour bénéficier aux EPCI ayant intégré un SAN au fil des réformes territoriales, puisque, vous le savez, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, votée par votre assemblée, a supprimé le statut de syndicat d'agglomération nouvelle au 1 janvier 2017, ce dernier ayant d'ailleurs disparu dans les faits au 1 janvier 2016. Ainsi, le Gouvernement a souhaité maintenir les droits existants des SAN, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, en prenant une disposition en loi de finances pour 2016 qui vise les fusions des communautés d'agglomération elles-mêmes issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle. Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité, à compter de l'année 2013, étendre cette modalité dérogatoire de calcul de la richesse d'un territoire aux dotations de péréquation horizontale, qui, je le rappelle, ont été augmentées de manière inédite durant le quinquennat. Ainsi, pour le calcul des contributions et reversements au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, le potentiel fiscal agrégé de l'ensemble intercommunal issu d'un SAN est pondéré pour la part du potentiel fiscal correspondant à ce dernier, dans l'objectif de poursuivre l'accompagnement de ces collectivités aux caractéristiques et charges particulières, telles que je viens de les décrire. À l'occasion des débats parlementaires sur la loi de finances rectificative pour 2016, un amendement, examiné à l'Assemblée nationale et repris par le Sénat, visait à restreindre l'application de la pondération du potentiel fiscal à la seule cotisation foncière des entreprises, la CFE. Le dépôt tardif de cet amendement, quelques heures avant qu'il ne soit discuté, n'a logiquement pas rendu possible la réalisation d'une étude d'impact et n'a donc pas permis d'en apprécier les effets sur les finances des collectivités concernées. Cela nous interroge d'ailleurs sur le processus de fabrique de la loi, l'évaluation des dispositions adoptées devant y prendre une place encore le Gouvernement a néanmoins émis un avis de sagesse, considérant que l'amendement n'avait pas d'impact sur les équilibres budgétaires de l'État et qu'il avait été présenté par ses auteurs comme plus conforme à l'intention du législateur que la mesure de maintien du régime dérogatoire votée en loi de finances initiale pour 2016. Le Gouvernement est aujourd'hui appelé à se prononcer sur cette proposition de loi relative au calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération, qui vise à rétablir la disposition initiale dans son champ initial, considérant après analyse que l'amendement voté en loi de finances rectificative produit des effets trop importants pour ces territoires. Le Gouvernement est favorable à cette proposition de loi, son adoption permettant d'éviter une rupture brutale, parce que non anticipée, des règles fiscales et financières, qui modifient de façon substantielle les conditions d'élaboration des budgets des intercommunalités concernées. Vous connaissez, comme moi, la demande pressante et légitime des élus à disposer d'un cadre financier et fiscal stable, tout comme leur exigence, également légitime, d'une association en amont de leurs représentants aux décisions qui les concernent et de simulations de ces dernières. Toutefois, j'entends les arguments selon lesquels la minoration du potentiel fiscal de ces territoires a mécaniquement des conséquences sur les autres territoires, tant les dispositifs sont imbriqués. Je suis attentive à ces remarques, dictées par le souci d'une répartition plus juste et plus solidaire des dotations.

en 2012 à 1 milliard d'euros en 2017, rend nécessaire de regarder précisément les critères qui déterminent les contributions de chacun, puisque moins contribuer pour les uns revient à plus contribuer ou moins percevoir pour les autres. Avec la disparition des syndicats d'agglomération nouvelle et leur intégration dans des EPCI de droit commun, il ne peut être fait l'impasse sur la question du retour, pour ces collectivités, à l'application du droit commun. Mais, parallélisme des formes, ce retour au droit commun des anciens SAN et de leurs EPCI actuels ne peut s'envisager, s'il devait l'être après analyse de l'adéquation des modalités de calcul de leur potentiel fiscal à leur richesse, que de manière progressive.

tend à repousser en 2018 la désignation des parlementaires membres des commissions DETR- dotation d'équipement des territoires ruraux -afin de tenir compte du renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du renouvellement partiel du Sénat en 2017 et de ne pas freiner les processus d'attribution de cette dotation,

aux spécificités des territoires couverts par les ex- SAN, tout en permettant par ailleurs de garantir le bon fonctionnement des commissions DETR, qui sont appelées à se réunir très prochainement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable au vote conforme de ce texte, pour lequel a été décidée la procédure d'examen accéléré,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui concerne les « villes nouvelles », mises en place dans les années 70, principalement en Île-de-France. s'étaient immédiatement organisées en intercommunalités, sous la forme principalement de syndicats d'agglomération nouvelle, ou SAN. Cette catégorie d'EPCI était temporaire, les SAN étant appelés à se transformer en EPCI de droit commun, et notamment en communautés d'agglomération. Dès 1999, il a été choisi d'accorder un avantage aux anciens SAN dans les modalités de calcul de leur potentiel fiscal, afin de tenir compte de leur niveau d'endettement particulièrement élevé, qui s'expliquait par les investissements considérables Depuis cette date, leur potentiel fiscal est divisé par deux environ, ce qui leur permet de recevoir une dotation d'intercommunalité plus importante. Cet avantage a été étendu en 2013 au potentiel fiscal agrégé, utilisé pour répartir le Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, ou FPIC. Indirectement, le coefficient s'est donc également appliqué au potentiel fiscal des communes membres de l'EPCI, compris dans le potentiel fiscal Lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2016, sur l'initiative de sa rapporteure générale, l'Assemblée nationale a diminué l'avantage accordé aux communautés d'agglomération issues de SAN. La présente proposition de loi vise à revenir sur cet article, en s'appuyant sur deux arguments. D'une part, l'amendement était passé inaperçu à l'Assemblée nationale, ayant été présenté comme la « correction d'une erreur ». D'autre part, les conséquences financières sont considérables pour les collectivités territoriales concernées, qui ne sont pas en mesure de les absorber en une seule année. Par ailleurs, les auteurs du texte reconnaissent qu'il pourra être nécessaire d'étudier si cet avantage est encore justifié aujourd'hui. Je rappelle que, à l'automne dernier, nous avions confirmé

La proposition de loi a été modifiée en séance : dans la version transmise, l'avantage est bien maintenu en 2017 dans les mêmes conditions qu'en 2016, mais il sera totalement supprimé à partir de 2018. En d'autres termes, pour l'après-2017, le dispositif retenu va plus loin que le texte adopté à l'automne. J'en viens aux conséquences financières. Nous n'avons pas pu obtenir de simulation pour ce qui concerne l'article adopté cet automne. En tout état de cause, il conduit à une baisse de la dotation d'intercommunalité perçue par ces EPCI et à une dégradation de leur solde au titre du FPIC. D'après les auteurs de la proposition de loi, les pertes seraient concentrées sur le FPIC et s'élèveraient à 26 millions d'euros en 2017. Ces montants représentent entre 3,2 % et 8,5 % des recettes réelles de fonctionnement des communautés d'agglomération concernées. Ces chiffres peuvent être comparés à la contribution au redressement des finances publiques, la CRFP, des communes, qui représente pour sa part environ 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement : la suppression du dispositif aurait donc effectivement des conséquences importantes

de le supprimer dans des conditions qui ne soient pas trop brutales. Le texte qui nous est transmis permet d'atteindre ces objectifs, dans la mesure où le dispositif disparaîtra en 2018, si rien n'est fait.

Je tiens à le souligner, la situation économique et financière a changé depuis 1999 : dans un contexte de baisse des dotations et de montée en puissance de la péréquation, les avantages accordés à des collectivités qui disposent de bases fiscales importantes sont plus difficiles à accepter. Néanmoins, l'importance des conséquences financières et le fait que le maintien de l'avantage est limité à 2017 ont conduit la commission des finances à adopter cet article sans modification. le souligne également, cette position est liée aux autres articles de la proposition de loi. Sa seule chance d'être définitivement adoptée avant la fin de la session est que nous l'adoptions conforme dès la première lecture. Or il me semble que l'article 2 apporte des précisions utiles : il repousse à 2018 la présence des parlementaires dans les commissions départementales de la DETR dans les seuls départements comptant plus de quatre parlementaires, en raison des difficultés pratiques à les désigner, à quelques mois du renouvellement de l'Assemblée nationale et du renouvellement partiel du Sénat. Enfin, je vous ai déjà présenté l'article 3, qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la pertinence de conserver le mécanisme dérogatoire de calcul du potentiel fiscal

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous étudions aujourd'hui une proposition de loi adoptée par nos collègues de l'Assemblée nationale relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des communautés d'agglomération issues de la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle. Ce texte vise à supprimer une disposition de la loi de finances rectificative pour 2016 promulguée voilà un peu plus d'un mois. Les syndicats d'agglomération nouvelle ont été créés en 1983 pour administrer les villes nouvelles, avec notamment pour mission de construire des logements et d'aménager des équipements d'accueil. Une fois ces missions menées à bien, les SAN ont dû se transformer en communautés d'agglomération. En contrepartie des investissements à réaliser, ces SAN, puis les communautés d'agglomération qui ont pris la suite, bénéficient depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, d'un régime de calcul du potentiel fiscal dérogatoire aboutissant à une dotation d'intercommunalité plus favorable. La loi de finances pour 2013 a étendu cette pondération aux ensembles intercommunaux pour déterminer l'attribution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, Cette fiscalité dérogatoire bénéficie aujourd'hui à six communautés d'agglomération et une métropole, par le biais de l'application au calcul du potentiel fiscal agrégé d'un coefficient dont résulte une pondération particulièrement importante, ayant des effets non négligeables sur leur dotation d'intercommunalité et le FPIC. L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 a remis en cause pour partie ce régime dérogatoire, en diminuant l'avantage accordé à ces communautés d'agglomération, par la réduction du périmètre de la pondération à la seule cotisation foncière des entreprises.

prévoit de restaurer ce régime dérogatoire des communautés d'agglomération issues de SAN, alors que les avantages dont elles bénéficient ne se justifient plus, vingt ans après leur mise en place et, surtout, dans l'état actuel de nos finances publiques. Concernant la première dérogation, relative au calcul du potentiel fiscal pour la dotation d'intercommunalité, c'est tout le potentiel fiscal des anciens SAN qui se trouve pondéré. Si, en 1999,

de l'extension de la dérogation au potentiel financier agrégé utilisée pour le FPIC, plusieurs remarques s'imposent. Le coefficient de pondération a permis à ces anciens SAN des participations au FPIC moindres de plusieurs millions d'euros. Malheureusement, la charge de la contribution est reportée sur les autres ensembles intercommunaux. L'absence de contribution de certains territoires doit être palliée par d'autres territoires, qui sont pourtant dans des situations financières tout aussi tendues, ce qui conduit à nous interroger sur les effets péréquateurs du FPIC.

Il avait été déclaré irrecevable, alors que l'amendement gouvernemental introduit à l'Assemblée nationale sur les commissions DETR me paraît avoir un lien tout aussi indirect avec le texte d'origine. Je me devais de le signaler. dirai que les dérogations dont bénéficient les anciens SAN créent une charge supportée injustement par les autres territoires, sans que cela soit justifié, et ce dans un contexte de contrainte financière. C'est la raison pour laquelle les membres du groupe du RDSE voteront à une très large majorité contre la présente proposition de loi. La parole

mais de mon point de vue utilement, avec la loi de finances rectificative de 2016, voilà moins de deux mois. Où est la cohérence ? Où est la lisibilité de l'action publique ? l'action publique ? Certes, le dispositif de minoration du potentiel fiscal, qui permettait aux communautés d'agglomération issues des syndicats d'agglomération nouvelle de bénéficier d'une DGF majorée, était justifié

Quand les syndicats d'agglomération nouvelle ont été introduits à partir de 1984, ils avaient pour mission d'accompagner le développement des villes nouvelles. Pour ce faire, ces neuf syndicats, créés dans la grande couronne parisienne et la région de Marseille, avaient besoin de dispositifs financiers adaptés. Ils devaient en effet faire face à de lourdes charges, notamment pour la création des infrastructures nécessaires à leur développement.

la DGF, afin de faciliter la transition des syndicats d'agglomération nouvelle vers un statut de communauté d'agglomération, était justifiée. Je trouve beaucoup plus discutable que, pour ces agglomérations, il ait été décidé en 2013 d'appliquer le potentiel fiscal minoré au calcul du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, créé l'année précédente. Ce potentiel fiscal pondéré s'établit aujourd'hui, je le rappelle, à près de la moitié du potentiel fiscal réel. Cela signifie que la richesse réelle de ces territoires est artificiellement minorée de moitié.

Je citerai trois raisons principales. La première, qui a été rappelée par Charles Guené, tient à la richesse fiscale de ces territoires. Leur développement, qui a nécessité de nouvelles infrastructures et des investissements lourds, a ensuite engendré des ressources qui en font aujourd'hui des territoires dont le potentiel fiscal est

Ainsi, désormais, l'attribution de moyens supplémentaires à une catégorie de collectivités se fait au détriment des autres collectivités. Troisième raison : dans le cadre de la réforme territoriale, la plupart des neuf communautés d'agglomération dont j'ai parlé tout à l'heure

Mes chers collègues, il ne s'agit pas d'opposer les territoires entre eux, comme on l'entend trop souvent ; chacun d'entre nous est attaché à son territoire et souhaite le voir se développer. C'est légitime. Mais, au-delà de cet attachement, je sais aussi que nous avons tous, ici, à coeur de veiller à la cohérence de l'action publique. Dans le traitement des territoires, le choix de l'équité doit inlassablement guider nos décisions. La parole

l'apparition de « villes nouvelles », dans les années 70, n'est pas le fruit d'initiatives locales. Bien au contraire, elle est le résultat d'un grand projet national d'aménagement du territoire.

Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après leur création, il ne semble pas moins illégitime d'envisager leur retour progressif dans le giron du droit commun. Une telle régularisation ne constituerait pas pour autant un abandon. Leur spécificité pourrait désormais être traitée non plus en référence à leur histoire, à leur création, mais sur la base de critères socio-économiques objectifs, que d'autres collectivités, malgré un passé différent, peuvent aussi bien satisfaire. Cette perspective de normalisation semble d'ailleurs unanimement partagée, y compris par les élus des collectivités locales Mais tel n'est pas l'objet de ce texte. Cette proposition de loi vise seulement à remédier, à titre conservatoire, aux conséquences indésirables d'un travail parlementaire sans

notre rapporteur général, à qui rien n'échappe, ... Eh oui ! ... a bien noté dans son rapport qu'en réalité la disposition n'était pas sans effet.

Je ne pense pas que ce dysfonctionnement législatif- je considère que c'en est un -soit le fait d'erreurs malencontreuses de tel ou tel parlementaire. Il me semble plutôt- mon collègue André Gattolin s'en est souvent fait l'écho à cette tribune -que nous observons là une conséquence concrète des problèmes structurels qui caractérisent l'examen automnal des textes budgétaires. Je voudrais en particulier pointer le détournement systématique du PLFR de fin d'année. dernier a pour seule vocation d'ajuster l'équilibre budgétaire de l'exercice qui s'achève par la prise en compte des aléas de gestion, il est en réalité utilisé comme une sorte de voiture-balai fiscale. Ajoutons à cela des délais très courts, vraiment très courts, et nous nous retrouvons, dans ce cadre, à examiner des mesures nombreuses, souvent complexes, dans un temps qui ne permet pas toujours un travail satisfaisant. Je pense d'ailleurs, monsieur le président, qu'il serait de la responsabilité du Sénat, compte tenu de l'attention particulière que nous portons à la qualité de la production législative, de conduire une réflexion approfondie à ce sujet. du cas qui nous occupe, à ce problème de procédure s'est ajoutée une difficulté, assez spécifique aux finances locales. En effet, lorsque l'on touche aux ressources des collectivités, quelle que soit la pertinence intellectuelle du mécanisme proposé, celui-ci doit doit toujours être évalué à l'aune de ses conséquences. Or la disposition du PLFR n'avait fait l'objet d'aucune évaluation. Il y a d'ailleurs de quoi s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui encore, les seules simulations dont nous disposons sont celles qui émanent des cabinets privés mandatés par les collectivités concernées. Que nous n'ayons donc pas légiféré dans des conditions satisfaisantes pourrait déjà suffire, me semble-t-il, à justifier notre soutien à cette proposition de loi.

Quoi qu'il en soit, la formulation de l'article 1 me semble de nature à lever les craintes. En effet, la révision complète de la dérogation, avant la fin de l'année, n'est pas un simple engagement politique ; elle sera, par ce texte, inscrite dans la loi. En conclusion, compte tenu des conditions contestables dans lesquelles l'amendement au PLFR a été adopté, de la mauvaise évaluation de ses conséquences et de la révision éclairée

; elle est raisonnablement technique, puisqu'elle concerne un régime fiscal dérogatoire en matière de dotation d'intercommunalité et de Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales,

relatives aux seuils démographiques des intercommunalités. Je connais bien cette situation ancienne et sa récente actualité : sur les sept communautés d'agglomération concernées par cette fiscalité dérogatoire, trois se trouvent totalement ou partiellement dans mon département d'élection, la Seine-et-Marne. coopération intercommunale, le dispositif fiscal dérogatoire prévoyait l'application d'un coefficient de pondération au calcul du potentiel fiscal agrégé desdits territoires, afin de prendre en compte leur endettement exceptionnellement important, lié à la nécessité de construire rapidement l'ensemble des infrastructures, des équipements publics et des logements, notamment sociaux, dans des proportions souvent très supérieures, pour ces derniers,

L'application d'une telle abrogation aurait un impact non négligeable pour les finances des EPCI concernés. À titre d'exemple, pour la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, la perte serait de près de 4 millions d'euros en 2017 et de 9 millions supplémentaires à l'horizon 2020

Or les villes nouvelles sont le fruit et le symbole d'une politique d'aménagement du territoire voulue par l'État. Elles ont largement contribué à urbaniser, à structurer et à développer des territoires, dans le cadre d'une démarche portée par les pouvoirs publics nationaux.

que d'activités structurantes, la logique étant celle, souhaitable, du développement polycentrique de la métropole parisienne et de son environnement périurbain. Il en est de même pour les territoires concernés situés aux portes des métropoles urbaines de province.

de logements par an à certaines périodes. Il a donc fallu élaborer des systèmes de soutien à l'investissement et aux charges nouvelles et accepter des niveaux d'endettement colossaux. Oui, mais l'activité économique accueillie fournit des ressources élevées », m'objecterez-vous. Certes ! Les potentiels fiscaux sont en effet élevés, mais cette richesse est trompeuse, puisque le niveau de la dette est exceptionnellement haut. Le remplacement de la fiscalité économique directe par des dotations d'État normées et stagnantes, sinon en baisse, annule les effets vertueux de la croissance, dont les territoires concernés ne bénéficient plus, qu'auparavant, alors que leurs charges afférentes à l'augmentation continue des populations et des services et équipements liés ne cessent de croître. Il nous revient donc, à nous, parlementaires, d'assurer à ces territoires, y compris sur le plan budgétaire, une sortie progressive d'un tel état d'exception. À l'heure où les élus recouvrent en partie leurs pleines capacités d'intervention, nous ne pouvons leur faire payer la facture d'un aménagement voulu à l'origine par l'État, lequel en assure aujourd'hui encore la maîtrise, puisqu'il accorde lui-même les permis de construire au titre des règles particulières des opérations dites d'intérêt national, C'est cette spécificité qui a justifié que nous, législateurs, adoptions des dispositifs particuliers pour ces territoires : urbanisation soutenue imposée, dispositions financières de soutien justifiées.

de dispositifs en sifflet : la loi Rocard de 1983 avait prévu un amortissement sur dix ans de l'harmonisation des taux de fiscalité entre les zones d'agglomération nouvelle, ZAN, et les territoires dits « hors ZAN Cette réflexion doit être conduite selon une entière concertation avec les territoires concernés, fondée sur une véritable étude d'impact, dans le cadre de la loi de finances, et non pas au détour d'un amendement de dernière minute à un projet de loi de finances rectificative. Le groupe socialiste votera en faveur de cette

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte dont nous discutons aujourd'hui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 2 février dernier,

permettre l'étude indispensable de la mesure proposée et de sa portée et faciliter le travail des rapporteurs respectifs des deux assemblées, celui du Sénat préconisant même l'adoption conforme du texte voté au Palais-Bourbon. D'autres propositions de loi attendent toujours dans la navette parlementaire et n'ont pas encore trouvé le chemin de l'ordre du jour.

du jour. La grande aventure des villes nouvelles, ce projet d'aménagement du territoire de la fin des Trente Glorieuses, voulu et pensé par le pouvoir au tournant des années 70, porté financièrement par la Caisse des dépôts et consignations, s'est achevée il y a quelques années par la dissolution des syndicats d'agglomération nouvelle mis en place, sur chaque territoire, pour définir les outils de la croissance et du développement. Là où se trouvaient, le plus souvent, des noyaux urbains anciens, isolés au sein d'ensembles ruraux plus consistants, nous avons assisté à l'émergence de nouvelles villes, d'infrastructures collectives, de services, de routes, de voies ferrées et de ponts, de gares, d'équipements publics,

Dans le département du Val-d'Oise, depuis 1975, sur dix nouveaux habitants, près de quatre sont venus résider dans l'une des communes de la nouvelle. En Essonne se sont développées deux villes nouvelles, l'une autour de la ville devenue préfecture et qui s'appelait Évry-Petit-Bourg, l'autre entre Corbeil et Melun, dans le périmètre de la ville nouvelle de Melun-Sénart.

Sud Seine-Essonne-Sénart. La dissolution des syndicats a en effet entraîné une recomposition des territoires. En Essonne, ce qui fut Évry s'est regroupé avec Corbeil, et a fini par se joindre à Melun-Sénart, par-delà les limites départementales, ce qui fait de notre nouvelle communauté d'agglomération un ensemble tripolaire autour d'Évry, de Corbeil et, dans une moindre mesure, de Savigny-le-Temple. de Grigny et de Ris-Orangis, qui sont confrontées aux problématiques des politiques urbaines, et nous obtenons la raison profonde qui provoque l'examen du texte qui nous occupe. n'est lui-même pas immobile. Pendant que les villes nouvelles s'achèvent et se découvrent de nouveaux problèmes, le paysage des finances locales évolue.

Évidemment, le développement économique des villes nouvelles a fait de ces territoires des contributeurs nets potentiels du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. La réforme de la carte intercommunale par le biais des lois MAPTAM et NOTRe a rendu la facture, aujourd'hui, particulièrement salée. Lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale a été pointé le montant des contributions exigibles,

En effet, la charge de la péréquation dite horizontale, entre EPCI à fiscalité propre, alors que le nombre des EPCI diminue, revient en définitive de plus en plus cher.

notamment à certaines villes à caractère industriel ancien et à population modeste, qui sont, dans les faits, pénalisées d'avoir su conserver leurs activités économiques et leur caractère populaire, y compris aux portes de la capitale. La question de fond posée par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est bel et bien celle du devenir de la péréquation, ce principe introduit dans notre Constitution, et celle du sens que la loi doit lui donner. Mes chers collègues, lorsqu'un fonds de 1 milliard d'euros, soit 2 % environ des recettes fiscales des collectivités locales, commence à poser problème en raison de sa conception « horizontale », il importe de se demander si la péréquation ne doit pas retrouver le sens de la verticalité et bénéficier d'une ressource dédiée, définie au niveau national. Au-delà du débat d'aujourd'hui, c'est bien de cela qu'il s'agit : de la justice fiscale et financière, au service du strict intérêt des populations, seule véritable motivation de toute péréquation. Notre groupe est très réservé sur l'équité d'une telle mesure au regard de la situation d'autres communes qui connaissent des difficultés équivalentes, et souhaite en outre manifester

cette proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale il y a quinze petits jours et adoptée par nos collègues députés voilà tout juste une semaine, revient sur les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016, adoptée en décembre dernier.

Cet article minore l'avantage accordé aux communautés d'agglomération comportant un ancien syndicat d'agglomération nouvelle, ou SAN, pour les modalités de calcul de leur potentiel fiscal.

La loi de finances pour 2013 a étendu l'application de ce coefficient au potentiel fiscal agrégé- ce dernier entre en ligne de compte dans les modalités de contribution au FPIC -des ensembles intercommunaux constitués d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un SAN et de ses communes Les mouvements en cours de fusion d'EPCI auraient pu cependant faire perdre à ces territoires le bénéfice de cette pondération. En conséquence, l'article 157 de la loi de finances pour 2016 prévoyait que cette pondération bénéficie également aux communautés d'agglomération issues de la fusion d'EPCI dont l'un au moins était un SAN s'étant transformé en communauté d'agglomération avant le 1 janvier 2015. L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 a remis en cause ce dispositif de manière précipitée, en minorant l'avantage accordé à ces communautés d'agglomération.

La pondération du potentiel fiscal des communautés d'agglomération comportant un ancien SAN a toujours porté sur l'ensemble du potentiel fiscal, et non sur les seules bases de CFE.

pour Paris-Vallée de la Marne, dont 3,8 millions dès 2017. La présente proposition de loi vise donc à éviter ces pertes de recettes considérables et brutales, par un retour à la situation antérieure, dans l'attente d'un nouveau dispositif, que nous serons bien obligés d'adopter, avec une sortie en sifflet, ce qui est généralement ce

Je lis partout, et constate souvent, que les délais pour légiférer sont trop longs. En l'occurrence, une proposition de loi déposée le 2 février- je dis bien le 2 février -sur le bureau de l'Assemblée nationale pourrait, aujourd'hui, 16 février, être votée conforme ! Quel talent, et quel démenti cinglant à tous ceux qui se plaignent d'une prétendue lenteur de la procédure législative

Comme cela a déjà été exposé par notre rapporteur, l'excellent Charles Guené, avec quelques difficultés malgré tout, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a pour objet de revenir sur les dispositions d'un amendement voté dans le cadre du PLFR pour 2016 et visant à modifier les modalités de calcul des potentiels fiscaux des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle. L'amendement présenté par notre collègue députée Christine Pires Beaune tendait, à juste titre, d'une part, à limiter la pondération applicable au calcul du potentiel fiscal servant de base au calcul de la dotation d'intercommunalité et, d'autre part, à supprimer ce principe de pondération pour la répartition du FPIC.

Je me contenterai de commenter la seconde dérogation, qui porte sur le FPIC et qui a pour conséquence de transférer de l'ordre de 30 millions d'euros des territoires « ex-SAN » vers les autres territoires de notre pays. Si l'on peut comprendre une pondération du potentiel fiscal au moment de la transformation des SAN en communautés d'agglomération, on peut s'étonner qu'un amendement adopté en 2013 ait pu adapter cette pondération au calcul du potentiel financier agrégé de ces territoires, faisant des communautés contributrices au

qu'il conviendrait d'annuler aurait, s'il était maintenu, des effets financiers majeurs pour les territoires ex-SAN. Il est dommage que, parallèlement, personne n'ait jugé utile de se préoccuper de l'impact des changements de périmètres sur les montants de FPIC mis à la charge des autres territoires.

situation impose une nouvelle réflexion sur la manière dont nous délibérons sur des dispositifs financiers qui ont des conséquences majeures.

La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Je mets aux voix l'article 1.

En plus de la perte de ressources que cette réforme a entraînée pour le bloc communal, les communes et intercommunalités ont été sollicitées pour organiser entre elles la solidarité au travers du Fonds national au point que le gel, en 2017, du montant de ce fonds apparaît aujourd'hui comme le résultat de la mobilisation des élus. C'est dire combien ce qui se passe avec les villes nouvelles est intéressant, mais ne saurait être déconnecté de l'ensemble des difficultés que connaissent les communes. Il convient donc de s'interroger sur le devenir des modes de péréquation des ressources entre collectivités territoriales. La sensible réduction des rentrées fiscales liée à la disparition de la taxe professionnelle appelle en effet d'autres mesures que celle conçue en 2012, qui renvoie les élus locaux et les territoires les uns contre les autres, sans considération réelle pour la situation des populations. Aucun dispositif horizontal ne sera parfaitement satisfaisant. Dès lors, la nécessité d'une péréquation verticale se pose. Cette solution doit, à nos yeux, être privilégiée. Voilà ce que nous attendons du rapport prévu à l'article 3 du présent texte. C'est pourquoi nous proposons d'élargir son périmètre à l'ensemble des collectivités territoriales et des EPCI. Nous attendons également de ce rapport la production de simulations.

commission ? Cet amendement vise à modifier le champ du rapport demandé au Gouvernement, qui concernerait alors l'ensemble des collectivités territoriales et non plus les seuls anciens SAN.

Je vais vous donner un exemple pour essayer de vous convaincre de nos bonnes intentions, mes chers collègues. La Seine-et-Marne a été victime d'inondations en juin dernier.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

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique

abouti à une conclusion positive. J'en suis heureux. C'était prévisible en raison de l'excellent climat qui a prévalu à l'occasion de l'examen de ce texte,

par les députés. De même, l'essentiel des ajouts votés par l'Assemblée nationale ont recueilli l'accord des sénateurs membres de la commission mixte paritaire. Les divergences de fond, peu nombreuses, ont porté sur trois points l'extension aux polices municipales du nouveau cadre d'usage des armes, le champ des procédures ouvrant droit au bénéfice des dispositions relatives à l'anonymat et la question de l'intervention des agents de l'administration pénitentiaire aux abords immédiats des établissements. Ces divergences ont pu être surmontées grâce à un esprit de large consensus républicain, qui doit s'imposer sur ces questions, surtout dans le contexte actuel.

tout en validant le dispositif retenu par le Sénat afin que les éventuels recours devant la juridiction administrative soient purgés dans des délais raisonnables, la commission mixte paritaire a retenu le système voté par les députés tendant à rendre obligatoire, en cas d'avis négatif rendu par l'autorité administrative et en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement du salarié dont le comportement

ne fasse plus référence aux abords immédiats des établissements, car cela rend inopérantes les dispositions pour les établissements pénitentiaires situés en zone urbaine. Là encore, comme pour l'interruption du périple meurtrier,

des élus locaux pour apprécier leurs besoins ! Quoi qu'il en soit, cet assouplissement va dans le bon sens. Nous avons également validé l'accès des parties au dossier de la procédure devant la chambre de l'instruction, le rétablissement du délit en cas de « parloir sauvage » avec des personnes détenues,

hier, les députés ont adopté le projet de loi relatif à la sécurité publique tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire. Je m'en réjouis moi aussi, tout comme je me suis réjoui de l'adoption de ce texte en première lecture par le Sénat le 24 janvier dernier. D'une manière générale, ce projet de loi, qui a recueilli une large majorité au sein des deux chambres, est le résultat d'un débat constructif, apaisé et marqué par le sens de l'intérêt général. À cet égard, je veux d'emblée remercier le rapporteur, François Grosdidier,

même si un certain nombre de divergences ont pu être exprimées. Encore une fois, je veux souligner l'esprit républicain qui a prévalu lors de l'examen du projet de loi, ici, au Sénat, comme à l'Assemblée

aux difficultés croissantes d'exercice du métier de policier, de gendarme et, plus généralement, de dépositaire de l'autorité publique, dans un contexte où la violence qui prend pour cible les représentants de l'État a désormais franchi un palier que nul ne saurait contester.

inédites menées au sein de la police et de la gendarmerie et qui inclura plusieurs mesures concernant le management et la reconnaissance du travail accompli. Je rendrai ces mesures publiques le 27 février prochain,

tous tenus. C'est ainsi que nous répondrons aux difficultés auxquelles les forces de l'ordre sont confrontées au quotidien. C'est ainsi que nous leur apporterons la confiance, la reconnaissance, la sérénité qu'elles méritent et dont elles ont besoin pour accomplir leur devoir de façon plus apaisée. À cet égard, vous comprendrez

À Aulnay-sous-Bois, des actes d'une gravité et d'une violence aussi intolérables qu'exceptionnelles ont été commis sur un jeune homme par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Ces actes, je les ai immédiatement condamnés ; les quatre policiers incriminés ont été immédiatement suspendus. La justice a été saisie, et il lui revient- et à elle seule -d'établir très clairement et sans aucune ambiguïté les conditions de l'interpellation qui a donné lieu à ces actes inacceptables, ainsi que de qualifier ces actes. Je veux de nouveau rappeler, avec solennité et gravité, le devoir d'exemplarité qui doit guider l'action des forces de sécurité, même et surtout lorsque la force et la contrainte légitimes doivent être employées. C'est dans le rapport respectueux entre la population et les forces de l'ordre que notre pacte républicain puise, et doit puiser, sa force. Il n'y a pas d'alternative. Cela signifie que les forces de l'ordre doivent être exemplaires et irréprochables, et tout comportement qui n'obéit pas aux règles de l'éthique et de la déontologie est sanctionné.

et de jeter l'opprobre sur toute une institution, pilier de la République. Il y a aujourd'hui près de 250 000 membres des forces de sécurité- police et gendarmerie -dans notre pays ; je pourrais y ajouter les effectifs de police municipale, qui agissent également dans le respect total de l'État de droit.

Je veux souligner les six axes qui structurent ce texte. Le premier est la modernisation et l'unification du cadre d'usage des armes guidées par les principes dégagés par la jurisprudence. Je n'y reviens pas, si ce n'est pour indiquer que l'application du 1° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure aux agents de police municipale est, je crois, un point final satisfaisant pour tout le monde. Le deuxième axe est la protection accrue des dépositaires de l'autorité publique au travers de la préservation de leur identité, et ce dans des conditions strictes et sous le contrôle des autorités judiciaires saisies des procédures. L'ultime version de l'article 2 concilie parfaitement, selon moi, les différentes exigences qui devaient être prises en compte. Le troisième axe est le renforcement des peines pour certaines atteintes à l'autorité publique

dans un souci de complémentarité avec les forces de sécurité intérieure. Enfin, le sixième axe est la complémentarité accrue des différents acteurs de la sécurité, avec le souci permanent de ne jamais induire de confusion dans les rôles

les sénateurs, je veux de nouveau me féliciter de l'esprit de rassemblement et de consensus avec lequel nous avons oeuvré collectivement sur ce projet de loi. Ce faisant, nous avons contribué à garantir et à sanctuariser ce que j'appelle « le socle de sécurité » nécessaire à notre

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis le début de la vague d'attentats que connaît notre pays, les forces de sécurité sont chaque jour mises à rude épreuve. Particulièrement exposés, certains policiers l'ont payé de leur vie ; je pense aux deux agents de la police nationale à Magnanville, le 13 juin 2016, ou encore à Clarissa Jean-Philippe, policière municipale à Montrouge, tuée en 2015 par Amedy Coulibaly. Dans ce contexte de menace terroriste sans précédent dans notre pays, il était indispensable de s'interroger sur le régime juridique de l'usage des armes par les forces de sécurité, non seulement par les policiers et les gendarmes, mais aussi par les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle. Bien entendu, la question de l'usage des armes face à cette menace terroriste sans précédent devait être revue. Pour autant, dans notre République, il ne saurait être question d'envisager un usage plus laxiste, d'abandonner nos principes de droit il faut à la fois permettre aux forces de l'ordre de se défendre- c'est évident -et respecter les règles que nous nous sommes fixées, qu'elles soient d'ordre constitutionnel ou conventionnel. La réflexion sur ce sujet a été marquée, cela a été rappelé, par deux rapports importants : celui de M. Guyomar, en juillet 2012, mais surtout celui de Mme Cazaux-Charles, rendu en novembre 2016. Leur analyse est convergente. Tous deux regrettent, d'une part, l'absence de lisibilité de ce régime d'usage des armes et, d'autre part, l'absence de cadre commun et spécifique aux policiers et aux gendarmes. Soumis à de fortes pressions, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale doivent, dans le feu de l'action, prendre des décisions extrêmement rapides dont les conséquences peuvent avoir de fortes répercussions. Cette réalité est parfois tragiquement mise en lumière par l'actualité. Notre législation devait donc évoluer afin de renforcer leur protection et de clarifier certaines situations dans lesquelles l'imprécision des textes est une source de confusion pour les agents comme pour les juges. Les régimes d'usage des armes sont aujourd'hui trop hétérogènes. Les agents de la police nationale sont soumis aux dispositions de droit commun fixées par le code pénal concernant la légitime défense. Sur le papier, le papier, le régime dont bénéficient les militaires de la gendarmerie nationale est plus large. Il est défini par le code de la défense, qui reprend les dispositions d'un décret de 1903, elles-mêmes héritées du XIX siècle Ces dispositions leur permettent d'employer la force armée lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux. On est donc loin de la légitime défense applicable aux policiers Récemment, le législateur a amorcé une évolution avec la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. Cette loi a autorisé les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national à faire usage de leur arme en cas d'« absolue nécessité », s'ils sont confrontés à un « périple meurtrier », afin de prévenir tout risque de réitération lors d'une tuerie de masse. On nous propose aujourd'hui d'aller un peu plus loin, ou plutôt, on nous propose de regarder le régime des armes dans sa globalité et de le faire évoluer de manière unifiée et cohérente. Cette évolution, dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, nous paraît opportune et raisonnable. Nous espérons qu'elle s'accompagnera d'une formation renforcée à l'usage des armes de nos forces de sécurité et d'un entraînement régulier, qui est son corollaire indispensable. Les dispositions indispensable. Les dispositions relatives à la protection de l'anonymat des agents intervenant dans les procédures pénales et douanières prévues à l'article 2 nous paraissent nécessaires dans la mesure où il s'agit, encore une fois, d'assurer à nos agents la protection à laquelle ils ont droit dans le cadre de leur mission. Je voudrais profiter de mon intervention pour évoquer un article passé un peu plus inaperçu, introduit à la faveur d'un amendement du député Gosselin l'article 10 , qui vise à relancer l'expérimentation d'un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales, tel que prévu par la loi du 9 juillet 2010. Monsieur le ministre, je vous ai écrit à ce sujet en décembre dernier, ainsi qu'à Mme Laurence Rossignol. Ma saisine reste sans réponse à ce jour, un oubli Il me paraît en effet intéressant de reprendre cette expérimentation qui, dans la pratique, n'a pas pu être réellement testée comme cela était initialement prévu. Si je regrette que le périmètre proposé dans l'article 10 reste identique à celui adopté en 2010, je souhaite que cette fois-ci, vraiment avoir lieu sur le terrain. Le système proposé le mérite : il correspond au type de protection demandé par les victimes, à savoir celui visant à empêcher leurs agresseurs de s'approcher d'elles. Des pays voisins l'ont mis en place avec un réel taux de réussite. d'oeuvrer après promulgation de ce texte à sa mise en place opérationnelle. Par ailleurs, notre groupe se réjouit que la disposition visant à réduire le nombre d'assesseurs siégeant à la cour d'assises spéciale ait été confirmée par veux dire un mot sur le délit de consultation de sites internet djihadistes. Le Conseil constitutionnel a censuré la semaine dernière une disposition que nous avions introduite dans la loi du 3 juin 2016. Vous le savez, l'opportunité de créer un tel délit est débattue au Sénat et à l'Assemblée nationale de manière régulière depuis 2012. Je me félicite que la commission mixte paritaire nous ait permis de réintroduire ce dispositif que j'estime indispensable. Chacun sait ici le type de propagande que l'on peut trouver sur ces sites. Leur toxicité n'est plus à démontrer. Nous ne pouvons pas nous contenter de savoir que ces écrits sont une composante d'autres incriminations pénales nous devons punir le simple fait de consulter régulièrement ces sites, sauf lorsque l'on s'aperçoit que cette consultation est le fait d'un journaliste, d'un chercheur. Le dispositif

constitue un cadre indispensable pour protéger les agents qui sont chargés d'assurer la sécurité de nos concitoyens au quotidien, mission d'autant plus périlleuse du fait de la menace terroriste qui pèse sur notre pays. La parole

nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre du projet de loi, tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire, relatif à la sécurité publique. L'examen de ce texte, qui constitue la réponse législative du Gouvernement à la mobilisation des policiers à la suite de l'attaque de Viry-Châtillon, en Essonne, intervient dans un contexte particulier que nul ne peut ignorer. Il y a quinze jours, Théo, vingt-deux ans, a été gravement blessé lors d'une opération de contrôle à Aulnay-sous-Bois. Il affirme avoir été victime d'insultes racistes, de coups et avoir subi un viol. Hospitalisé, opéré en urgence, il s'est vu prescrire soixante jours d'incapacité totale de travail. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ces faits terribles ne doivent pas être utilisés pour jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession, sur ces hommes et ces femmes dévoués à leur tâche et qui font parfois l'objet, on l'a vu, d'attaques d'une violence inouïe. Toutefois, l'affaire Théo et les répercussions qu'elle a eues dans toute la société doivent nous interroger. Avons-nous oeuvré, en tant qu'hommes et femmes politiques, en tant que législateur, à protéger nos concitoyens des violences policières ? Avons-nous pris des mesures efficaces pour restaurer la confiance brisée entre la population et sa police ? Le constat est plutôt négatif, et notre responsabilité collective est, je crois, engagée. Les attentats, le tout-sécuritaire réclamé sur bien des bancs de l'Assemblée nationale et des travées du Sénat, ont abouti à une interdiction de parler de certaines défaillances chez nos forces de l'ordre, à un véritable tabou. Qui aura tenté de rappeler la nécessité d'un récépissé pour les contrôles d'identité, ce que nous avons fait ici aux côtés de nos collègues communistes ? Qui aura plaidé pour le retour d'une véritable police de proximité ? Qui aura réclamé plus de transparence de l'usage des armes par les forces de sécurité ? Ceux qui l'ont fait ont été accusés, parfois avec outrance, d'avoir osé exprimer de la défiance envers des forces de l'ordre dont l'unique objectif serait de nous protéger des terroristes.

Nous parlons aujourd'hui d'encadrer les circonstances dans lesquelles les policiers pourront utiliser leurs armes et de l'usage que police et gendarmerie font de la force publique dont ils sont dépositaires. Dans un tel contexte, la première des choses est de s'atteler, me semble-t-il, à faire la lumière sur un certain nombre d'éléments. C'est un des combats que mène l'ONG ACAT France depuis des années. Ainsi, pendant dix-huit mois, ACAT a réalisé un état des lieux des violences policières en France. Au terme de son enquête, elle a publié un rapport intitulé pour briser le silence autour de cette question. Ce rapport, qui repose sur l'analyse de quatre-vingt-neuf cas d'utilisation excessive de la force par la police et la gendarmerie, met en évidence dans quelles conditions, avec quelles méthodes et quelles armes sont commises les violences policières. Au regard du bilan humain découlant de l'utilisation de certaines armes, Flash-Ball et Taser notamment, et des gestes d'immobilisation, c'est probablement leur usage qui devrait être réformé et encadré plus strictement. Ce rapport met également en évidence la relative impunité dont bénéficient les forces de l'ordre puisque, sur les quatre-vingt-neuf situations examinées, seules six ont fait l'objet de condamnations au jour de sa conclusion. Comme le résume très bien le rapport, « difficulté de déposer plainte, d'obtenir une enquête effective, disparition d'éléments probants, déclarations manifestement mensongères des forces de l'ordre, durée excessive des procédures pénales, menace de condamnation pour outrage et rébellion Obtenir justice est souvent un parcours du combattant. Lorsque les agents sont condamnés, les sanctions sont faibles au regard d'autres condamnations pénales prononcées en France. Les images de l'arrestation de Théo, les constatations médicales surtout et son témoignage ont empêché les habituelles contestations des faits et remises en question de la personnalité de la victime. Beaucoup doit être fait pour endiguer les phénomènes violents de part et d'autre ainsi que pour restaurer la confiance entre police et population. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui ne nous semble être ni un facteur d'apaisement ni la garantie d'une protection des forces de sécurité comme des citoyens.

que la procédure législative a été concomitante à de graves affaires : Viry-Châtillon, Carrousel du Louvre, Aulnay-sous-Bois.

dans l'exercice de leurs missions était absolument nécessaire et très attendue par les personnels de police qui sont- tous les orateurs l'ont dit -extrêmement sollicités dans le contexte lié aux attentats et exposés à des risques croissants et de plus en plus violents. Le projet de loi est une réponse à la demande légitime de protection exprimée par les fonctionnaires de police. Il concerne plusieurs volets, notamment l'usage des armes par les forces de l'ordre et la protection de l'identité des enquêteurs. Ces évolutions juridiques prennent tout leur sens

humains et matériels des forces de police de notre pays. Je le rappelle, le plan de sécurité annoncé par le Gouvernement le 26 octobre dernier

pour alimenter notre réflexion sur l'examen du texte. Je tiens à souligner l'équilibre des dispositions obtenues lors du débat parlementaire ainsi que la qualité

Comme le Conseil d'État le précisait dans son avis sur le projet de loi, l'alignement du cadre d'usage des armes pour toutes les forces de l'ordre de l'État est tout à fait justifié par le rapprochement des conditions d'intervention des policiers, gendarmes, douaniers et militaires sur le terrain. Les forces de police et de gendarmerie sont de plus en plus mobilisées pour des opérations de sécurité

toutes les garanties exigées par les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, notamment celles qui sont relatives aux conditions d'absolue nécessité et de proportionnalité. L'article décrit d'ailleurs précisément

La mission d'information sur les polices municipales menée en 2012 avec mon collègue François Pillet a permis d'appréhender la diversité des territoires. Tenant compte de réalités locales diversifiées,

est arrêtée par le maire. Nous avons largement débattu de cette question. L'armement apparaît nécessaire lorsque les policiers municipaux interviennent ponctuellement comme forces supplétives de la police ou de la gendarmerie. Cette condition doit

permettre aux policiers municipaux affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle de procéder à des palpations de sécurité. C'est un progrès

délictuelles a été conservé. De plus, la commission mixte paritaire a ouvert la possibilité pour l'agent de bénéficier des dispositions relatives à l'anonymat pour des délits punis de moins de trois ans d'emprisonnement lorsque, en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Ce dispositif

nationale, qui est à l'origine de la première, a proposé des ajustements à la loi de 1955 sur l'état d'urgence, notamment sur les modalités d'assignation à résidence, l'information du parquet et l'alignement des horaires de perquisitions administratives

terroristes ou en faisant l'apologie, disposition qui a été censurée le 10 février dernier par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une

en conformité bien évidemment avec les préconisations du Conseil constitutionnel, cette disposition. Enfin, notre groupe voudrait saluer une disposition passée

après l'accord trouvé en commission mixte paritaire viennent donc les conclusions de ce projet de loi, dont l'examen expéditif nous laisse songeurs tant les dispositions qu'il comporte sont lourdes de conséquences. Dicté par la grogne policière de l'automne dernier, à la suite de l'agression violente que nous avons condamnée, comme toutes les autres d'ailleurs, de quatre fonctionnaires à Viry-Châtillon, ce texte nous est soumis à quelques mois de la fin de la législature, dans un contexte préélectoral et de menace terroriste qui pose plusieurs questions, dont celle de son opportunité. Désormais, avec l'entrée en vigueur des dispositions de ce texte, les policiers pourront ouvrir le feu dans cinq situations jusque-là réservées aux gendarmes face à la menace de personnes armées ; lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ; lorsqu'une personne cherche à échapper à leur garde, qu'ils ne peuvent l'arrêter autrement et qu'elle présente une menace lorsqu'ils ne peuvent arrêter autrement un véhicule en fuite présentant une menace ; la cinquième et dernière situation reprend la possibilité d'ouvrir le feu déjà prévue par la loi du 3 juin 2016 en cas de « périple meurtrier », c'est-à-dire dans le cas où un attentat vient d'être commis et que les personnes sont en cavale et susceptibles de tuer de nouveau. Comme nous l'avons dit lors de l'examen du texte au Sénat le mois dernier, de nombreux syndicats, associations et professionnels du droit et de la sécurité ont dénoncé ce texte. Avant son examen par l'Assemblée nationale, la Ligue des droits de l'homme a appelé les députés à rejeter ce texte « qui autorise les forces de l'ordre à ouvrir le feu dans des conditions qui vont augmenter le risque de bavures Plus critique encore, le Syndicat de la magistrature estime que les forces de l'ordre « se considéreront légitimes à user de leurs armes, et potentiellement de tuer, dans des conditions absolument disproportionnées ». Nous estimons également que ce texte présente un danger, d'abord pour les policiers eux-mêmes. Car rappelons que, si le nouveau régime est adopté, il continuera à être soumis au respect des principes d'« absolue nécessité » et de « stricte proportionnalité », comme l'exige la convention européenne des droits de l'homme dans son article 2, qui consacre le droit à la vie. C'est pourquoi si l'exécutif pense qu'il est nécessaire de légiférer pour libérer les coups de feu, il oublie que l'Europe a déjà condamné à plusieurs reprises des gendarmes ayant fait usage de leur arme « illégitimement Ainsi, dans deux avis distincts, le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'inquiètent du risque pour les policiers de croire, à tort, à une plus grande liberté.

sur le malaise des policiers rendu public en janvier- je vous invite à le lire -, elle dénonce « une fausse bonne mesure parce qu'au fil du temps une jurisprudence de plus en plus restrictive a vidé de son sens l'article 2338-3 du code de la défense sur lequel se fonde la légitime défense applicable aux gendarmes Définitivement, la loi n'est pas le moyen adapté face au malaise policier ! Trois autres mesures contenues dans le texte suscitent notre inquiétude. Tout d'abord, les dispositions concernant l'anonymisation des enquêteurs dans les actes de procédure portant sur un crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement remettent en question le respect du contradictoire et l'exercice des droits de la défense. Nous partageons la position de la Ligue des droits de l'homme sur le sujet le principe d'une police anonyme n'est pas acceptable en démocratie, sauf à en faire un corps étranger à la Nation. Ensuite, comme de nombreuses autres mesures ajoutées par la droite sénatoriale, le renforcement des prérogatives des policiers municipaux en matière de sécurité publique a été retenu. Nous y sommes fermement opposés. Rappelons que la police municipale n'est pas placée sous la même autorité que les policiers nationaux et les gendarmes, elle n'exerce pas les mêmes missions et ne dispose pas des mêmes prérogatives. En outre, elle ne comporte pas de corps d'inspection. Enfin, et c'est une première dans l'histoire de la République, une disposition législative censurée par le Conseil constitutionnel le 10 février dernier a été réintroduite le 13 février suivant. Il s'agit du rétablissement dans le code pénal du délit de consultation habituelle de sites djihadistes, qui avait été créé par la loi antiterroriste du 3 juin 2016. Depuis 2012, nous sommes opposés à l'inscription dans la loi de ce délit dangereux pour le respect des droits fondamentaux, notamment la liberté d'information. Nous nous félicitions de la censure du Conseil constitutionnel et déplorons sa réinscription

en matière de sécurité sont tout autres. Je le répète, il est temps de restaurer une police de proximité soucieuse du vivre ensemble, dont tout le monde parle, dans le même temps des garde-fous pour éviter d'éventuelles dérives policières, en mettant en place par exemple- n'en déplaise à certains -les récépissés lors des contrôles d'identité. nous constatons, une fois encore, et je le dis avec une certaine gravité, que ce gouvernement n'aura fait que partager la vision du tout-sécuritaire propre aux politiques de sécurité publique les moins progressistes. Vous l'aurez compris, nous voterons contre ce texte, ce qui signifie qu'il n'y a pas de consensus. Le consensus, mes chers collègues, ne peut se résumer à un accord entre le parti socialiste et la droite ! Très bien

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis janvier 2015, en raison de leur engagement aux avant-postes dans la lutte contre le terrorisme, les 270 000 personnes qui constituent nos forces de l'ordre sont exposées à un risque particulier, supérieur à celui qu'elles connaissent en temps normal. Plusieurs attaques, comme celle qui a eu lieu très récemment contre des militaires de l'opération Sentinelle déployés dans l'enceinte du Carrousel du Louvre à Paris, permettent de caractériser ce risque spécifique. Nul ne peut le contester. Dans ces conditions, il est nécessaire de réfléchir à de nouvelles méthodes et à de nouveaux dispositifs pour améliorer les conditions de travail et l'efficacité de nos forces de l'ordre, en veillant tout particulièrement à réduire leur vulnérabilité à de futures attaques terroristes. C'est l'esprit du projet de loi qui nous a été soumis par le Gouvernement, dont la finalité nous semble tout à fait justifiée. À ce stade des discussions, dans le cadre d'une procédure accélérée, que l'on peut regretter compte tenu de l'importance des mesures proposées et du périmètre des personnes concernées, l'examen des solutions proposées nous rend cependant plus circonspects. En effet, la première revendication des agents de la police nationale porte sur le régime de l'utilisation de leurs armes à feu et sur la légitime défense. Cette préoccupation comporte en réalité deux questions qu'il faut traiter de manière distincte d'une part, la question de la sécurité juridique de l'utilisation des armes pendant le service et, d'autre part, la question de la vulnérabilité des agents des forces de l'ordre en dehors de leur service ainsi que la protection de leur famille. concerne la vulnérabilité des agents en dehors de leur service et de leur famille, un problème manifeste comme l'a tristement illustré le double assassinat de Magnanville, notre attention doit être toute particulière. Nous ne pouvons tolérer que des agents publics et leurs familles soient victimes de telles menaces en raison du service qu'ils rendent à la Nation. De ce point de vue, la possibilité pour les agents

nous contestons l'idée que l'augmentation du quantum des peines pour outrage et rébellion, également proposée, puisse affaiblir le sentiment de vulnérabilité des forces de l'ordre.

À l'avenir, les solutions visant à restaurer la confiance entre ces différents acteurs, entre les parties prenantes, devraient au contraire être recherchées dans le cadre d'une lutte contre des perceptions qui ne sont pas toujours justement fondées. De la même manière, nous ne sommes pas convaincus par l'utilité de la réforme proposée du régime d'utilisation des armes. Il est vrai que ce projet de loi de loi uniformise les régimes s'appliquant aux gendarmes et aux policiers, ce qui permettra au moins de lutter, là aussi, contre des perceptions prégnantes. Pour autant, comme le soulignent des organisations professionnelles de magistrats, le nouveau régime ne permettra pas de lever toute l'impression diffuse d'insécurité juridique qui dissuade parfois nos agents de faire usage de leur arme.

Il est vrai qu'il est « dangereux de laisser penser que les forces de l'ordre pourront faire un usage plus large de leurs armes ». En réalité, les mêmes contraintes et le même régime de responsabilité D'autres solutions pourraient être recherchées pour permettre une utilisation plus sereine des armes à feu par les forces de l'ordre : une augmentation des moyens accordés à la formation au maniement des armes ou la concentration des moyens de formation sur des brigades spécialisées seules habilitées à porter des armes, comme cela se fait au Royaume-Uni. Une réflexion pourrait également s'ouvrir sur une éventuelle réforme du régime de responsabilité pour les dommages résultant de l'usage d'armes à feu. Malheureusement, la procédure accélérée ne nous a pas permis d'étudier toutes les options envisageables permettant de répondre plus efficacement à ces attentes qui sont, je le répète, légitimes. Au contraire, nos discussions se sont dirigées sur des sujets plus éloignés des préoccupations de nos forces de l'ordre. Pour toutes ces raisons, les membres du RDSE ont très majoritairement fait le choix de l'abstention sur ce projet de loi relatif à la sécurité publique.